Cet amendement vise à porter de six mois à un an le délai pendant lequel les défauts de conformité apparus sont présumés exister au moment de la délivrance d'un bien d'occasion. L'objectif est de renforcer la confiance des consommateurs dans les biens d'occasion, donc d'inciter au réemploi. L'idée me semble intéressante, mais il faut veiller aux équilibres de la relation entre vendeur et acheteur, comme pour les autres propositions relatives à la garantie légale de conformité. En outre, ayons à l'esprit que cela risquerait de conduire à une augmentation du prix des produits d'occasion. La commission demande l'avis du Gouvernement sur cet amendement.

Nous souhaitons faire de la garantie légale de conformité un outil au service de l'allongement de la durée de vie des produits et de la transition vers une économie circulaire. Pour ce faire, il faut réparer plutôt qu'échanger. Or certains

Ce taux tombe à 20 % pour les produits hors garantie. Un produit hors garantie est donc peu susceptible de faire l'objet d'une réparation. De plus, pour certains matériels, le remplacement par un produit neuf est relativement fréquent. C'est le cas pour les appareils de petit électroménager, mais aussi les téléphones portables, les petits équipements électroniques ou encore les tablettes numériques.

recyclées. Nous l'avons déjà dit, étendre la durée de vie des produits est le moyen le plus efficace, non seulement pour endiguer la production de déchets, mais aussi pour favoriser la préservation des ressources. C'est dans cette optique que nous proposons de créer, comme le préconisent l'association Halte

Cette disposition, qui existe dans de nombreux pays européens, permet à la fois de mieux protéger les consommateurs contre les pannes prématurées et d'inciter les vendeurs à réparer plutôt qu'à échanger les produits, dans le cadre de la garantie légale de conformité, pour économiser les coûts que représente le traitement de pannes potentielles.

de ces amendements, nous attirons toutefois leur attention sur la portée limitée de la notion de priorité, qui n'est d'ailleurs pas prévue dans la directive de 1999. En outre, la rédaction proposée écrase des dispositions indispensables à la mise en oeuvre de la garantie, en précisant les modalités selon lesquelles le vendeur arbitre en fonction de la demande

En outre, cela pourrait conduire à des stratégies d'acheteurs visant à demander de donner la priorité au remplacement, y compris dans des cas où le vendeur n'aurait pas le choix, pour des raisons de coût. La commission a donc émis un avis défavorable

La garantie légale de conformité est un dispositif qui permet, à partir de l'achat du bien, de disposer d'une protection juridique en cas de défauts initiaux du produit, pour une durée fixée lors de l'achat initial ; cela constitue donc un contrat entre le vendeur et l'acheteur.

Actuellement, une fois la garantie expirée, l'usager peut faire le choix de se tourner vers un réparateur professionnel, mais si, à la suite d'une réparation, une défaillance intervient, le consommateur n'est plus couvert par aucune protection juridique. Cette incertitude et le coût dissuadent largement de recourir à cette solution. Un nombre croissant de réparateurs offrent déjà une garantie de trois mois à leurs clients à l'issue de la réparation. Nous souhaitons encourager et encadrer cette pratique. Nous proposons donc d'allonger la garantie légale à six mois à compter de la réparation du produit. en 2016 par l'association 60 millions de consommateurs, 92 % des Français sont convaincus que les produits high-tech et électroménagers sont volontairement conçus pour ne pas durer. Dès lors, on comprend mieux que, aux premiers signes de fatigue et de bogue d'un appareil, quand la date de fin de garantie approche, la plupart des consommateurs préfèrent en racheter un neuf.

de l'économie circulaire. Cette pratique favorise l'emploi local et de proximité et contribue, de ce fait, à l'aménagement du territoire. C'est aussi un moyen efficace de diminution de l'empreinte écologique, grâce à l'allongement de durée de vie des produits, la fabrication étant la phase la plus polluante de celle-ci. Les enquêtes d'opinion le montrent, une large majorité des citoyens préféreraient faire réparer leurs appareils plutôt que de les renouveler, mais, aujourd'hui, dans 60

Mettre en place une garantie sur la réparation des biens serait un moyen efficace d'inciter le consommateur à faire réparer ses appareils. Cet amendement relève du même esprit que les deux précédents, mais il

à la suite d'une réparation, en vue de généraliser une pratique déjà mise en place par certains réparateurs et d'inciter à recourir davantage à la réparation, plutôt qu'au remplacement du produit. L'objectif semble intéressant. Toutefois, il s'agit d'une fausse bonne idée, car cela risque d'augmenter significativement le coût de la réparation. En outre, il ne paraît pas tout à fait cohérent de rendre tout réparateur responsable du bon fonctionnement de l'ensemble du produit lorsqu'il répare un de un de ses éléments, en particulier lorsque l'on connaît la structuration du secteur de la réparation, qui comprend de nombreux indépendants et beaucoup de petites entreprises. Cette contrainte risque de créer une entrave à la réparation, donc d'aller à rebours de l'objectif visé.

L'amendement a pour objet d'étendre à l'obsolescence programmée la définition de la tromperie commerciale inscrite dans le code de la consommation,

Il en est une qu'il conviendrait, à notre sens, d'intégrer dans la définition de celle-ci : l'introduction volontaire d'une défectuosité, d'une fragilité, d'un arrêt programmé ou prématuré,

programmée est définie comme le recours à des techniques par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d'un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie pour en augmenter le taux de remplacement. Elle constitue un délit puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 euros. La difficulté à appliquer cette disposition ne vient pas d'abord d'un problème de définition de son périmètre, car la notion de techniques permet déjà de couvrir un champ large. Le problème consiste plutôt à identifier le caractère intentionnel de la démarche en vue de réduire la durée de vie du produit.

relative à la mention que doit comprendre la facture des biens neufs en vue d'assurer une complète information du consommateur sur l'existence de la garantie légale de conformité. qui a été remis au Parlement en avril 2017 soulignait bien qu'elle est souvent méconnue du consommateur et qu'un certain nombre de commerces en profitent pour proposer des garanties commerciales payantes, dont l'intérêt est parfois limité par rapport à la garantie légale de conformité.

la méconnaissance de ce dispositif est bien identifiée et conduit parfois les consommateurs à opter pour des garanties commerciales payantes à l'intérêt limité par rapport à cette garantie légale gratuite. Il s'agit cependant d'un enjeu pour les distributeurs, qui auront peut-être à ajuster leurs systèmes de facturation.

À l'heure où les distributeurs disposent des moyens nécessaires pour enregistrer les achats, refuser d'appliquer la garantie sous prétexte que le client ne dispose plus de son ticket de caisse

Actuellement, lorsqu'un contrat est conclu par voie électronique, le professionnel est tenu de conserver ce contrat et d'en garantir l'accès aux consommateurs pendant une durée de dix ans à compter de sa conclusion. Cet Cet amendement vise à ce que le contrat soit conservé pendant toute la durée de la garantie légale de conformité du bien. Or je rappelle que la loi a prévu que celle-ci couvre les biens pendant une durée de deux ans suivant l'achat.

Cet amendement vise à imposer l'affichage de la durée de vie pour certains produits, en fixant comme critère une valeur supérieure à 30 % du salaire minimum interprofessionnel En raison des difficultés inhérentes à l'évaluation fiable de la durée de vie des produits, que nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer en commission, l'avis de la commission est défavorable. Sans parler de sa mise en oeuvre, qui serait très complexe, cette proposition va à l'encontre de l'approche retenue par le Gouvernement, qui entend développer l'affichage

L'amendement tend à demander au Gouvernement la remise d'un rapport sur l'opportunité de créer une plateforme numérique recensant la disponibilité des pièces détachées.

L'obsolescence logicielle est une forme insidieuse d'obsolescence programmée. Nous la rencontrons particulièrement dans notre quotidien avec nos smartphones, sur lesquels nous recevons régulièrement des demandes de mise à jour du logiciel d'exploitation. la pomme s'en est fait la spécialité ... Au fur et à mesure de ces mises à jour, notre téléphone devient plus lent, moins adapté aux nouvelles possibilités techniques offertes et, à terme, obsolète. Les industriels incitent ainsi les consommateurs à se procurer des téléphones plus modernes pour pouvoir profiter de la palette entière des fonctionnalités proposées. Si nous devons laisser aux industriels la possibilité d'améliorer leurs produits et d'offrir des améliorations en temps réel aux consommateurs, il faut cependant réfléchir à un encadrement strict de toute forme d'obsolescence logicielle qui rendrait les appareils inutilisables.

ne saurait connaître de vecteur plus efficace que notre jeunesse, et donc l'éducation. Nous connaissons l'argument selon lequel on attend trop de l'école, cette dernière ne pouvant transmettre tous les savoirs et toutes les aptitudes. Nous l'entendons, mais

Nous le savons, c'est jeune que l'on apprend facilement, et ce sont les bonnes habitudes acquises dans la jeunesse qui sont les plus durables. C'est jeune que l'on se montre enthousiaste pour les activités manuelles.

vise à compléter la rédaction élaborée par la commission, qui prévoit « une sensibilisation à la réduction des déchets, au réemploi et au recyclage des produits et matériaux ainsi qu'au geste de tri ». Il semble pertinent d'intégrer également

constitue une dimension essentielle de la transition écologique. En initiant les collégiens au prolongement de la durée de vie des biens, on favorisera les comportements de consommation responsables pour le futur,

Cet amendement vise à récrire l'article 4 , introduit en commission, afin de remplacer une simple demande de rapport par un dispositif concret. Il s'agit de rendre obligatoire au 1 janvier 2021 l'installation d'un compteur d'usage sur les gros appareils ménagers et les équipements informatiques et de télécommunication.

Cela a été dit : de tels compteurs d'usage sont déjà en place sur un certain nombre de biens, mais ils ne sont pas visibles par le consommateur. Il s'agit, par cet amendement, d'en faire un outil permettant d'informer le consommateur sur la durée de vie

? Tous ces amendements visent à généraliser la mise en place d'un compteur d'usage sur certaines catégories d'équipements électriques et électroniques, à savoir les gros appareils ménagers et les équipements informatiques et de communication. Si la démarche est intéressante, elle ne saurait être généralisée sans recourir préalablement à des expérimentations. En outre, les produits concernés relèvent de marchés internationaux, ce qui semble peu compatible avec la prise d'une initiative strictement française, conçue comme une obligation.

dans un élan unanime ! L'article 70 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte définit un certain nombre d'orientations visant à lutter contre l'obsolescence programmée. Il prévoit un certain Il prévoit un certain nombre d'expérimentations en vue d'encourager des pratiques commerciales et industrielles plus vertueuses, dont l'une a trait à « l'affichage, sur la base du volontariat, de la durée de vie des produits afin de favoriser l'allongement de la durée d'usage des produits manufacturés grâce à l'information des consommateurs L'information des consommateurs est un facteur clé pour la réussite de la nécessaire transition écologique, parce qu'elle constitue l'une des premières étapes d'un changement des comportements. Si le concept d'obsolescence programmée n'a pas été retenu par le Gouvernement dans sa stratégie de communication, préférant l'effectivité des actions visant à promouvoir la réparabilité, il n'en reste pas moins qu'il s'agit là d'un fléau écologique pour la planète et financier pour les consommateurs. Il est temps de passer aux actes en actionnant tous les leviers déjà prévus, afin de mettre le pays en marche vers la réduction des déchets, le réemploi des objets et des matériaux et la nécessaire économie de la fonctionnalité, pour réussir la transition

en particulier sur le bilan des expérimentations prévues en matière d'information du consommateur sur la durée de vie des produits. En réalité, la remise d'un rapport sur le sujet était bien prévue par la loi de 2015, au plus tard pour le 1 janvier 2018. 2018. À ce jour, le Parlement n'en a pas été destinataire. Mme la secrétaire d'État pourra sans doute répondre sur ce point. En l'état, une demande de rapport est donc déjà prévue par le droit en vigueur.

L'industrie saura mettre sur le marché des produits durables, dans la mesure où on le lui impose, comme elle savait le faire par le passé : les célèbres machines à laver Vedette

importante dans la lutte contre l'obsolescence programmée, l'indice de durabilité est plus intéressant dans la mesure où il permet d'attirer l'attention de nos concitoyens sur des produits dont le cycle de vie est plus long, au-delà de leur réparabilité.

référence à des expérimentations relatives à l'affichage de la durée de vie des produits. En raison de difficultés techniques, liées en particulier à l'évaluation de la durée de vie et à la façon de présenter cette information au consommateur, les travaux de l'Ademe avaient été réorientés vers la réparabilité,

à polémiques de la part notamment d'une partie de l'industrie agroalimentaire, mais, en fin de compte, il est en voie de s'imposer, non seulement en France, mais aussi dans d'autres pays européens. Pour parvenir à mettre au point un indice de ce type, il faut du temps et de la concertation.

particulièrement du système d'exploitation, inadaptée à ses capacités techniques-puissance, stockage, mémoire vive. Par exemple, les vieux ordinateurs ne sont pas suffisamment puissants pour faire tourner les nouvelles versions de Windows. De la même manière, les vieux téléphones portables ne tolèrent pas toujours les mises à jour récentes de leur système d'exploitation. Dès lors, l'appareil périclite, notamment à cause de failles de sécurité qui ne sont plus corrigées. Une variante consiste en une mise à jour trop lourde pour la puissance de l'appareil, qui, du coup, fonctionne mal, voire plus du tout.

et 172 rectifié -ou installer un autre système d'exploitation sur la machine, tout particulièrement un logiciel tiers ou logiciel libre. Ces logiciels gratuits et en libre accès sont en général peu gourmands en mémoire et en puissance. Pour les ordinateurs, le plus connu d'entre eux est Linux. Pour les téléphones portables, le phénomène est plus récent, mais il se développe. certains appareils sont construits de sorte à ne pas autoriser l'installation d'un autre système d'exploitation que celui prévu par le fabricant. C'est le cas de certains ordinateurs et d'à peu près tous les modèles de téléphones portables.

Déjà examiné en commission, cet amendement vise à imposer des conditions vraiment spécifiques d'information du consommateur sur les mises à jour du système d'exploitation des appareils Définir un régime spécifique à ce sujet dans la législation française paraît avoir une portée limitée. Intervenir sur ces questions nécessiterait de mener un travail d'expertise spécifique, pour établir un état des lieux

ensuite à délivrer des mises à jour correctives pour chacune des mises à jour évolutives. Cela complexifierait énormément la gestion de ces logiciels. Quand bien même on la renverrait au décret,

vise à lutter contre l'obsolescence programmée et à allonger la durée de vie des produits en interdisant tout procédé technique visant à rendre irréparable ou non reconditionnable un produit.

qui sont des piliers de l'économie circulaire, en luttant contre des pratiques industrielles totalement opposées à l'économie circulaire. Entre 2014 et 2017, le volume des produits ménagers réemployés ou réutilisés a augmenté de 30 %. Selon certains sondages, les trois quarts des Européens préfèrent réparer réparer un appareil que le changer. Ce marché en pleine expansion et générateur d'emplois doit être soutenu. Il apparaît donc nécessaire de lutter contre toute technique industrielle visant à rendre un produit ou un bien irréparable ou non reconditionnable. La parole est à M.

pour présenter l'amendement n° 669 rectifié. Comme les précédents, cet amendement vise à interdire les techniques employées par certains fabricants pour programmer l'obsolescence des biens qu'ils fournissent. Nous le savons, c'est devenu un sport international : certains fabricants mettent en oeuvre des procédés qui rendent les biens qu'ils produisent absolument irréparables. C'est ce phénomène qui a amené la naissance de l'association Halte

Par exemple, les smartphones, ordinateurs ou tablettes numériques sont parfois conçus avec des composants collés ou soudés, ce qui empêche toute réparation, même par des professionnels.

ses caractéristiques essentielles. Ce n'est qu'en rendant possible dans tous les cas la réparation que nous pourrons en finir avec la culture de l'usage unique, du jetable, créer des emplois locaux dans ces filières et développer une véritable économie circulaire. J'y insiste, il

Ces amendements identiques portent sur un sujet connexe à l'obsolescence programmée, puisqu'ils visent à interdire les techniques, notamment en matière de logiciels, qui tendent à rendre la réparation ou le reconditionnement d'un appareil impossible hors circuits agréés.

Là encore, nous nous heurtons à d'importantes difficultés. D'abord, il n'est pas aisé de démontrer qu'une technique, surtout une technique logicielle, vise spécifiquement à empêcher la réparation hors des circuits agréés.

Elles déclenchent l'obsolescence prématurée des équipements, dès lors que le fabricant ou l'éditeur de logiciels le décide en forçant l'utilisateur à procéder à ces mises à jour. Il convient de distinguer les mises à jour correctives des mises à jour évolutives.

Le non-respect de cette obligation serait passible d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Je vous rappelle, mes chers collègues, que la problématique de l'obsolescence logicielle avait bien été identifiée par l'excellent rapport de la mission d'information sur l'inventaire et le

Il me semble que le niveau de contrainte que cela créerait pour les metteurs sur le marché serait particulièrement drastique. Je tiens à rappeler que le délit d'obsolescence programmée se caractérise par une volonté de tromperie du producteur, dont le but serait de raccourcir sciemment et de façon anormale la durée de vie des produits. La mesure proposée ici va au-delà de cette définition. Au surplus, une durée de dix ans serait en tout état de cause très longue par rapport à la durée de vie de ce type d'équipements. Il ne faut pas oublier que l'on parle ici d'appareils électroniques ou électroménagers.

Il est particulièrement insupportable qu'un appareil parfaitement fonctionnel soit rendu inutilisable par une simple mise à jour logicielle. Les pratiques des constructeurs de téléphones en la matière sont tout à fait déloyales et honteuses : elles ont d'ailleurs valu à Apple et à Samsung, en Italie, des amendes de 10 millions et 5 millions

pourrait même être cumulative dès lors que l'infraction serait constatée sur chaque produit issu d'une série de production. Or l'objectif de la loi me semble plutôt être de sanctionner des manquements systématiques et répétés aux nouvelles obligations qu'elle prescrit.

Il n'est pas pertinent de préciser que le manquement doit être répété pour être sanctionné. Il revient aux services de l'État d'apprécier l'importance du manquement et, le cas échéant, de le sanctionner en fonction des circonstances. À défaut, l'intégralité des régimes de sanction pourrait faire l'objet d'une telle précision, ce qui affaiblirait le droit de la consommation. J'ajoute que les contrôles en matière de consommation sont déjà suffisamment sporadiques pour ne pas ajouter une limitation supplémentaire au pouvoir des agents.

L'appréciation de la sanction, en particulier de son montant, en fonction du caractère répété ou non des manquements, appartient aux autorités de contrôle, sous

Cet amendement, déjà examiné en commission, vise à accroître les sanctions encourues en cas de manquement à l'obligation de fournir des pièces issues de l'économie circulaire pour certaines catégories d'équipements électriques et électroniques. Il s'agit d'une obligation nouvelle, pour laquelle il nous semble adapté adapté de reprendre un régime de sanctions existant, en l'occurrence celui qui est prévu pour l'obligation de même nature s'appliquant déjà au secteur automobile et dont s'inspire directement l'article 4 du projet de loi. La commission a par conséquent émis un avis défavorable

Par exemple, si 100 produits font l'objet d'un défaut d'information, l'amende peut aller jusqu'à 300 000 euros. Il me semble que les montants actuellement prévus dans le projet de loi sont proportionnés et suffisants, mais je m'en remettrai sur ce point à la sagesse de la Haute Assemblée. Je mets

essentiels de la chaîne de l'économie circulaire. Toutefois, les consommateurs et les responsables, professionnels ou particuliers, de la gestion initiale des déchets doivent également participer à l'effort de réduction de l'empreinte carbone. Cela passe d'abord par le tri,

La très grande majorité des membres du CNTE a soutenu cette mesure utile, qui participe de l'affirmation de la responsabilité environnementale des entreprises, notamment au regard de la santé au travail. Par ailleurs, la mise en oeuvre de cette disposition n'entraînerait aucun coût supplémentaire au regard des obligations existantes de fourniture d'informations concernant les installations classées, les contributions aux organismes à REP, la sécurité des consommateurs, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Nous espérons donc qu'une telle mesure pourra être adoptée. lorsqu'il est question des orientations stratégiques, de la situation économique ou de la politique sociale de l'entreprise. Le présent amendement vise, conformément à une recommandation du CNTE évoquée par M. Gontard, à instaurer un nouveau type de consultation sur les actions mises en place par les entreprises en matière d'économie circulaire et de gestion des déchets. En effet, si nous souhaitons réellement amorcer un virage en matière de réduction des déchets et de sensibilisation de la population à ces enjeux, nous devons agir à tous les niveaux et dans toutes les sphères.

Certes, prévoir une meilleure information des salariés sur les données et les réalisations de leur entreprise en matière d'économie circulaire est une bonne idée en soi, car cela permettrait de mieux les associer à la marche de l'entreprise et de les sensibiliser à cet enjeu.

En premier lieu, la rédaction actuelle permet déjà à une entreprise d'informer et de consulter les salariés sur ce point, car la gestion des déchets fait partie des questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise.

ce qui n'est pas le cas de la gestion des déchets. Il faut laisser aux entreprises la liberté d'associer leurs salariés sur cette question selon un mode plus souple que dans le cadre du CSE. Pour ces raisons, la commission a émis un avis défavorable

et d'alourdir encore les procédures de droit du travail collectif, qui sont déjà souvent jugées trop lourdes et contraignantes en France. L'information dont il est question ici

nous ne saurions nous satisfaire de ce progrès. Selon l'Ademe, chaque année, ce sont encore 10 millions de tonnes de denrées alimentaires qui sont gaspillées. Nous devons donc faire mieux et chercher où se trouvent nos marges de manoeuvre. Cet amendement vise ainsi à étendre l'un des dispositifs mis en place par la loi Garot de 2016, qui prévoyait que l'obligation de don aux associations d'aliments consommables, mais impropres à la vente par les centres commerciaux, ne concernait que les grandes et moyennes surfaces de plus de 400 mètres carrés. Cette mesure ayant permis de lutter activement contre le gaspillage alimentaire, il est proposé d'accroître son périmètre en permettant également aux centres commerciaux d'une surface inférieure à 400 mètres carrés de nouer des conventions de don avec les associations d'aide aux plus démunis. Quel

pour toutes les grandes et moyennes surfaces de plus de 400 mètres carrés, le conventionnement avec une ou des associations en vue de leur donner leurs invendus alimentaires. En réalité, rien n'interdit

les grands centres commerciaux, force est de constater que des progrès sont encore réalisables. Pour preuve, selon l'Ademe, 14 % des tonnages de nourritures gaspillées sont encore issus de la grande distribution. Bien que le code de l'environnement entérine le principe de la sanction, certains se refusent à jouer le jeu de la solidarité et préfèrent rendre certains aliments impropres à la consommation plutôt que d'en faire don aux associations d'aide aux plus démunis. En 2017, selon l'ONU, 820 millions de personnes au monde souffraient de sous-nutrition. Quand des hommes, des femmes et des enfants meurent encore de faim à notre époque, il est absolument intolérable que des géants commerciaux se permettent de gâcher volontairement de la nourriture. Afin de contrer ce phénomène bien réel en France, cet amendement vise à rendre les sanctions encourues plus dissuasives qu'elles ne le sont aujourd'hui. absence de conventionnement passerait d'une contravention forfaitaire de troisième classe à une amende de cinquième classe, et la sanction pécuniaire pour destruction de denrées alimentaires consommables serait portée de 3 750 euros 750 euros à 10 000 euros. Nous espérons que ces mesures permettront de mettre fin à l'impunité des acteurs de la distribution alimentaire, qui doivent participer à l'effort national contre la malnutrition et le gaspillage. Quel

qui ne respecteraient pas l'obligation de conventionner avec une association pour le don de leurs invendus alimentaires, et une amende de 3 750 euros pour les distributeurs du secteur alimentaire qui rendent délibérément impropres à la consommation des invendus alimentaires encore consommables.

jetés. Plusieurs initiatives ont été prises par le législateur, mais également par les associations, afin de contribuer à faire évoluer les pratiques. Les associations récupèrent des denrées alimentaires et les redistribuent à des particuliers se trouvant en situation de précarité. précarité. Au regard des enjeux écologiques, économiques et sociaux liés au gaspillage alimentaire, il est urgent de lutter contre ce gâchis en développant au maximum le don, la transformation ou la valorisation

caritatives la cession à titre gratuit des denrées alimentaires ne pouvant donner lieu à transformation ou à valorisation, avant qu'elles ne soient impropres à la consommation humaine. Le non-respect de cette obligation serait sanctionné. Ces dispositions entreraient en vigueur à partir du 1 janvier 2021. Quel l'avis de la commission ? Depuis la loi du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire, les commerces de détail alimentaires dont la surface de vente dépasse 400 mètres carrés ont l'obligation de proposer à une ou plusieurs associations habilitées de conclure une convention relative au don de leurs denrées alimentaires invendues.

Toutefois, il me semble qu'il fait porter une contrainte très forte sur des commerçants qui, considérés individuellement, ne vendent qu'un volume limité de denrées et n'ont donc pas les mêmes moyens que les commerces de détail et les grandes surfaces sur lesquels une telle obligation pèse déjà. Au demeurant, je remarque que de nombreuses initiatives ont été développées dans notre commune pour récupérer les invendus à la fin des marchés et les redistribuer gratuitement.

ainsi libellé : La parole est à Mme Esther Benbassa. Depuis plusieurs années, les dates limites de consommation appliquées par les industriels sur leurs produits frais ou secs connaissent d'importantes modifications, dans un sens favorable au au combat contre le gaspillage alimentaire. Certaines dates ont été supprimées pour des produits jugés non périssables, comme le sel ou le vinaigre, et d'autres ont été allongées, notamment pour les produits frais,

Les produits concernés sont les boîtes de conserve hermétiques et en bon état, les produits lyophilisés, les pâtes, le riz, les flocons d'avoine, les huiles, le miel et les épices. Cette proposition va dans le sens des règlements européens, qui encouragent vivement les États membres de l'Union européenne à lutter contre le gaspillage alimentaire, en supprimant des dates de péremption qui n'ont pas lieu d'être. À l'instar de nombreux produits vendus en vrac, par définition sans date de durabilité minimale, il convient, pour certains produits

De manière plus précise, c'est l'annexe X au règlement n° 1169-2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, d'application directe, qui fixe cette liste

si je partage votre objectif de clarifier l'information des consommateurs sur les dates de durabilité minimale des produits alimentaires, une interdiction simple n'est pas conforme au droit européen actuel. droit européen actuel. C'est pourquoi j'ai décidé d'agir à l'échelon européen pour modifier la mention d'information des consommateurs sur cette date, pour que celle-ci ne soit plus interprétée comme une échéance limite de consommation.

Il s'agit d'encourager l'éco-conception des produits et de responsabiliser les producteurs de produits non recyclables. En commission, la rapporteure a indiqué qu'il était préférable d'avoir recours à un dispositif d'éco-modulation

Par ailleurs, il apparaît que les éco-modulations ne s'appliqueront qu'aux produits soumis à une REP, alors que la présente taxe s'appliquera à tous les produits non recyclables, soumis ou non à une REP.

pour orienter les acteurs économiques vers des modes de production plus vertueux, car il s'agit là d'une logique punitive. À l'inverse, les éco-modulations déplafonnées par le projet de loi permettent de responsabiliser une filière de production et de créer un chaînage vertueux entre ses acteurs afin de les inciter à trouver de meilleures solutions. Les éco-modulations sont préférables aux taxations à plusieurs égards. D'une part, elles sont supportées par les producteurs et non par les consommateurs ; d'autre part, elles sont neutres pour le budget de l'État et peuvent directement financer des bonus sur les produits plus vertueux,

Je vous laisse imaginer les conséquences pour beaucoup de Français. En outre, si la notion de recyclabilité est très bien encadrée dans les filières REP, comme vous l'avez souligné, monsieur le sénateur, elle ne fait l'objet d'aucune définition

il serait intéressant d'examiner le traitement réservé aux denrées consommables saisies aux frontières, notamment dans les aéroports, par les services de l'administration douanière. Depuis un arrêté du 4 mars 2013, il est proposé aux douaniers de faire don aux associations des aliments saisis. Six ans après la publication de cet arrêté, il est temps d'en évaluer les

leur traitement, afin de quantifier la part consommable annuellement perdue dans les poubelles de nos administrations.

L'article 5 crée une obligation en priorité de réemploi ou de réutilisation, puis de recyclage, de produits neufs, pour les ventes directes comme pour les ventes en ligne. Tous les produits seront donc concernés, sans exception, sauf bien sûr ceux qui sont périssables ou dangereux pour l'environnement ou la santé humaine. Des sanctions financières seront prévues contre ceux qui ne respecteraient pas ces mesures anti-gaspillage ; des contrôles seront effectués par les services de l'État. L'objectif de la mesure est clair : encourager le don de qualité des grandes surfaces. Il s'agit de réduire le déficit chronique de certaines associations, notamment en produits d'hygiène. Interdire la destruction des invendus textiles permettrait d'économiser 250 000 tonnes de CO2 par an, soit l'équivalent des émissions de 125 000 voitures.

des dates limites de consommation. L'objectif est bien évidemment d'éviter la mise au rebut de produits qui seraient encore consommables, mais qui sont jetés en raison des dates affichées.

: La parole est à M. Éric Gold. La loi Garot relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire prévoit les conditions dans lesquelles les commerces de grande distribution cèdent leurs invendus alimentaires à une association d'aide aux plus démunis. Cette loi pionnière a entraîné une forte augmentation des dons de produits alimentaires aux associations caritatives. Si le bien-fondé de cette mesure ne doit bien sûr pas être remis en question, certaines de ses conséquences doivent être prises en considération par les pouvoirs publics. Les collectivités territoriales constatent en effet une augmentation significative des déchets alimentaires que les associations n'ont pas été en mesure de distribuer à leurs bénéficiaires. La gestion de ce nouveau flux de déchets incombe donc aujourd'hui aux collectivités. L'objet de cet amendement est de prévoir, dès la signature des conventions entre distributeurs et associations, les modalités de prise en charge de ces déchets. Il tend ainsi à préciser que la grande distribution est tenue de financer ou de pourvoir à la gestion des déchets issus des dons effectués aux associations. Les trois

seront signataires de la convention de dons de produits alimentaires entre distributeurs et associations. En effet, l'obligation de don des invendus alimentaires introduite

le dispositif ne traite pas aujourd'hui de la gestion des déchets suscités par les invendus alimentaires qui n'ont pas pu être redistribués par les associations aux bénéficiaires. Or les associations sont difficilement en mesure de refuser les dons proposés par la grande distribution, y compris lorsque les denrées en question sont impossibles à distribuer, soit parce qu'elles sont endommagées, soit parce que leur date limite de consommation ces denrées ne sont pas redistribuées, elles sont jetées par les associations et finissent dans le circuit de gestion des déchets ménagers. Leur gestion est donc assurée par le service public de gestion des déchets par le contribuable local, alors qu'il s'agit initialement de déchets d'activité économique produits par les distributeurs du secteur alimentaire, lesquels sont tenus de les gérer. Le dispositif en vigueur permet donc à un distributeur de donner aux associations des denrées qui sont sur le point de devenir des déchets, dont il aurait dû assurer le traitement, et de bénéficier en contrepartie d'une réduction d'impôts

Les collectivités territoriales constatent un afflux de plus en plus important de déchets issus des denrées alimentaires données aux associations n'ayant pas pu être redistribuées. Cet amendement vise donc à associer les collectivités à l'élaboration

En l'état, la commission craint que cet amendement premièrement ne jette le discrédit sur l'ensemble des distributeurs, alors que, dans l'immense majorité des cas, les choses se passent plutôt bien deuxièmement qu'il ne renverse le problème. Supposons ainsi qu'une association ne parvienne pas à écouler ses stocks, alors même qu'ils ont été remis en bon état : pour quelle raison reviendrait-il au distributeur de prendre en charge leur gestion comme déchets ? Nous allons, je pense, au-devant de multiples conflits.

entre les acteurs de la grande distribution et les associations concernant les dons de denrées alimentaires. Les auteurs de ces amendements pointent en effet une réelle limite du système actuel, qui peut conduire certaines grandes surfaces peu scrupuleuses à écouler des produits en les donnant à des associations,

5 prévoyant un contrôle aléatoire par les services de l'État de la qualité des denrées données. Associer toutes les collectivités concernées à toutes les conventions qui lient chaque grande ou moyenne surface à une association risque d'alourdir considérablement le système, sans pour autant apporter une bonne réponse.

des dons alimentaires. Or la loi Égalim d'octobre 2018 a déjà introduit l'obligation pour les distributeurs d'assurer la qualité du don. Un récent décret en précise les modalités d'application. De plus, les dispositions de la loi Garot, renforcées par la loi Égalim, prévoient un régime de sanctions en cas de non-respect des obligations de don alimentaire par les distributeurs. il n'apparaît pas utile de préciser dans la loi que l'État procède à des contrôles de ces dispositions. La loi le prévoit déjà. C'est pourquoi le Gouvernement propose de supprimer l'alinéa 2 de l'article 5.

ne s'appliqueraient pas « aussi longtemps que les conditions nécessaires pour réaliser le réemploi, la réutilisation et le recyclage ne permettent pas d'y procéder de façon satisfaisante au regard de l'objectif de développement durable.

la nécessité de hiérarchiser la gestion des déchets, en favorisant en priorité le réemploi, la réutilisation, puis le recyclage. L'amendement vise cet objectif en répondant à une demande très forte de la part des acteurs incontournables que sont les associations caritatives mentionner précisément le mot « don » dans le projet de loi. Il tend ainsi à favoriser la démarche solidaire du projet de loi en introduisant le don comme une solution prioritaire comprise dans le réemploi pour aider les personnes en situation de grande précarité.

Mme Catherine Dumas. La disposition de l'alinéa 4 de l'article 5, si elle n'était pas complétée, comme le prévoit cet amendement, pourrait favoriser la constitution de réseaux parallèles de distribution de certains produits dans des conditions illégales. En effet, l'instauration d'un ordre de priorité dans les modes de gestion des invendus est susceptible de produire des difficultés, notamment d'ordre juridique. Les produits issus d'un mode de distribution sélectif ou exclusif doivent le plus souvent faire l'objet de dégriffes avant de pouvoir être redistribués dans les réseaux associatifs et solidaires, afin de ne pas alimenter des réseaux parallèles de distribution. Or, comme vous le savez, cela n'est pas toujours possible. Je pense aux imprimés textiles portant des marques, des signes distinctifs, à certains types de chaussures ou éléments d'accessoires de mode tels que les fermoirs, les boucles. Cet amendement donc que l'obligation de suivi d'un tel ordre de priorité doit se faire dans le respect des principes du code de commerce, mais aussi et surtout dans celui des réseaux de distribution sélective ou exclusive.

Nous soutenons bien évidemment cette mesure importante, mais nous souhaitons, par cet amendement, proposer une précision importante. Il s'agit de faire du don aux associations agréées une possibilité supplémentaire au réemploi, à la réutilisation et au recyclage, afin de sortir de la situation ubuesque consistant à privilégier le recyclage ou la destruction d'un bien neuf et fonctionnel à son utilisation. Le meilleur déchet étant celui que l'on ne produit pas, il aura également un effet incitatif sur les quantités produites, les producteurs

destinés à la vente sont tenus de réemployer, de réutiliser ou de recycler leurs invendus. Il s'inscrit dans une démarche de lutte contre le gaspillage et de soutien à l'économie circulaire que nous soutenons, bien sûr. Afin de renforcer la portée de cette mesure, nous proposons, sur le même modèle que la loi Garot relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire, d'interdire de manière claire aux producteurs, importateurs ou distributeurs de détruire ou de rendre impropres au réemploi leurs produits neufs. Cet amendement vise à soutenir l'économie du réemploi, en garantissant, par cette précision utile, qu'elle sera la première sollicitée par des industriels qui pourraient, par facilité, vouloir se tourner en priorité vers le recyclage. Il s'agit par ailleurs d'une mesure de bon sens visant à éviter les comportements analogues à ceux que l'on a pu observer dans la grande distribution alimentaire.

Il nous semble sur le fond intéressant, puisqu'il est effectivement inconcevable d'imaginer la destruction pure et simple des invendus, comme le pratique par exemple Amazon.

soit d'abord le réemploi et en dernier lieu le recyclage. Nous partageons cette vision. Pour autant, nous restons quelque peu dubitatifs sur l'effet réel d'une telle mesure. En effet, le projet de loi organise de lourdes exceptions à cette obligation, notamment lorsque les conditions nécessaires pour réaliser le réemploi, la réutilisation ou le recyclage ne permettent pas d'y procéder de façon satisfaisante en fonction des objectifs de développement durable. Si l'affichage semble juste, la lettre de cette dérogation ouvre la voie à un contrôle selon nous incertain. Cette possible dérogation est extrêmement large, trop peu encadrée. Elle permettra au final à de nombreux producteurs de s'affranchir de l'obligation ainsi créée en ouvrant la porte à des dérives qui pourraient limiter les activités de réemploi et de réutilisation. Nous proposons donc purement et simplement de supprimer cette possibilité de dérogation qui nous semble mal formulée,

pour privilégier le réemploi, puis la réutilisation et à défaut le recyclage. En outre, la dérogation relative au développement durable permet d'intégrer des cas non couverts par la première dérogation relative aux risques fondés sur la santé ou la sécurité. Pour ces raisons, l'avis de la commission est défavorable

de commerce qui n'existe pas. Sur le fond, concernant les réseaux de distribution sélective, une telle restriction risquerait d'être exploitée par certains producteurs pour échapper complètement au dispositif de lutte contre les invendus. Pour des raisons de fond et de forme,

Les amendements n 161 rectifié et 257 rectifié visent à préciser que les entreprises ne peuvent délibérément rendre leurs invendus impropres au réemploi ou à la réutilisation, en reprenant une disposition analogue prévue pour la lutte pour la lutte contre le gaspillage alimentaire. Il existe une grande diversité de produits susceptibles de relever de ces invendus et l'interdiction de rendre impropres nous semble difficile à appliquer. L'avis de la commission est donc défavorable.

Cela étant, je retire l'amendement pour ne pas remettre en cause les avancées de la commission,

après l'alinéa 6 : « Parmi les invendus proposés par un producteur, un importateur ou un distributeur, les opérateurs de tri conventionnés par un éco-organisme au sens de l'article L. 541-10 du code de l'environnement et les associations et sociétés

? L'amendement n° 241 rectifié vise à empêcher les opérateurs de tri et les associations de l'économie sociale et solidaire de refuser des produits recyclables qui leur sont adressés par les producteurs ou distributeurs. Il n'existe pas de disposition analogue s'agissant de la lutte contre les invendus alimentaires. J'ajoute même que, à l'occasion de la loi Égalim, le législateur a précisé que les distributeurs de produits sont chargés de s'assurer de la qualité de leurs dons. Une telle proposition risque de faire des opérateurs du recyclage et des associations de l'économie solidaire des sortes de « poubelles » des grands acteurs de la distribution, sans capacité de refuser

non alimentaires s'applique aux plateformes de mise en relation de producteurs et d'acheteurs lorsqu'elles assurent la détention des produits. Autrement dit, il s'agit d'ajouter un critère de contrôle des stocks. C'est bien ainsi que le dispositif pourra effectivement s'appliquer. La commission a donc émis un avis favorable.

nous pensons qu'il appartient aux importateurs, aux producteurs et aux distributeurs de mettre en place des solutions pour le réemploi et le recyclage de leurs invendus, en passant le cas échéant des marchés avec les opérateurs de recyclage.

Je ne souscris pas non plus à votre proposition de faire peser l'obligation de traiter les invendus sur les opérateurs de recyclage, parce que ces importateurs et producteurs sont en contrat avec leur éco-organisme pour la gestion de leurs déchets. De plus, ce n'est pas parce qu'un opérateur de recyclage est conventionné par un éco-organisme qu'il est automatiquement en mesure de traiter l'ensemble des types de produits gérés par l'éco-organisme.

vis-à-vis des entreprises utilisatrices de leurs services. Seules les places de marché détentrices de produits invendus qui assurent une gestion logistique des produits pour leurs clients vendeurs seront soumises à l'interdiction d'élimination des invendus. Il s'agit d'une clarification utile à laquelle je suis favorable.

en cas de non-application de l'interdiction de destruction des invendus non alimentaires neufs prévue au présent article. Nous estimions en effet qu'une obligation non assortie de sanction n'en était pas vraiment une. vraiment une. L'adoption de l'amendement de la rapporteure a donc été une bonne chose. Toutefois, la solution retenue et les montants envisagés sont assez classiques et ne tiennent pas compte, selon nous, nous, de la spécificité du sujet qui nous occupe. Ainsi, il nous semble préférable de ne pas penser en termes de montant fixe de sanctions- 3 000 euros et 15 000 euros dans le cas présent -, mais en montant variable en fonction du prix de vente du produit bientôt illégalement détruit. nous estimons qu'il sera plus dissuasif d'appliquer une sanction proportionnelle au prix de vente- dix fois le prix, par exemple -plutôt qu'un montant fixe. À titre d'illustration, nous savons que cet article vise notamment les vêtements, particulièrement les vêtements de luxe. Appliquer une sanction de 15 000 euros sur un vêtement qui en coûte déjà plusieurs milliers ne serait pas nécessairement dissuasif, mais appliquer une sanction s'élevant à dix fois le prix de vente pourrait l'être davantage. Quel est l'avis de la commission ? La commission a déjà défini un régime de sanctions pour assurer l'effectivité de l'interdiction de destruction des invendus, en référence à un barème existant et connu en matière de droit de la consommation. Il ne nous paraît pas opportun de définir un système proportionnel au prix de vente des produits, qui complexifiera ce nouveau dispositif, dont la mise en place risque déjà quelque peu complexe. L'avis de la commission est défavorable. l'avis du Gouvernement ? Le régime de sanctions introduit par la commission sur l'aménagement et le développement durable me semble suffisamment dissuasif à ce stade. Ces sanctions financières seront mises en oeuvre dans les conditions du code de la consommation. Ainsi, si 100 produits n'ont pas été gérés conformément à l'interdiction d'élimination des invendus, la sanction encourue est de 100 fois 15 000 euros pour une personne morale, soit 1,5 million d'euros.

Nous savons que dans de nombreux cas les industriels ou les metteurs sur le marché préfèrent s'acquitter de sanctions financières, qu'ils peuvent assumer, plutôt que de changer leur méthode. En revanche, nous savons que ces mêmes personnes sont très frileuses à l'idée que leur image puisse être entachée par des pratiques peu vertueuses. peu vertueuses. C'est pourquoi nous proposons d'appliquer ce que certains appellent le au non-respect de destruction des produits non alimentaires neufs. Ces pratiques étant à l'opposé même du principe de l'économie circulaire et de la nécessaire lutte contre le gaspillage, nous devons mettre tout l'arsenal juridique possible en place pour y mettre un terme. Quel l'avis de la commission ? Au vu des préoccupations de la société civile vis-à-vis de la destruction des invendus, il nous paraît très pertinent d'ajouter une sanction complémentaire d'affichage ou de diffusion